La réforme défendue par Emmanuel Macron dans son programme présidentiel s'inspire notamment de la réforme fiscale suédoise de 1991 ayant instauré un impôt proportionnel de 30 % sur l'ensemble des revenus du capital. « La réforme du PFU [prélèvement forfaitaire unique] a été annoncée comme neutre budgétairement dans le programme présidentiel. Dans les faits, si la réforme n'engendre que des gagnants, son coût budgétaire pourrait être significatif. Notons qu'à l'heure actuelle le taux marginal d'imposition dans la deuxième tranche de l'impôt sur le revenu est de 14 %, auxquels s'ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux, soit un taux marginal total de 29,5 % pour les ménages aux taux marginaux les plus faibles ..., excepté pour les revenus d'assurance vie de plus de huit ans, le PFU constitue une diminution de taux par rapport aux taux des prélèvements libératoires déjà existants. Ainsi, selon notre évaluation, sur la base d'un PFU à 30 % avec possibilité de rester imposé au barème de l'impôt sur le revenu pour les ménages étant peu ou pas imposés, son coût budgétaire serait de l'ordre de 4 milliards d'euros. » Remercions les économistes de l'OFCE d'éclairer notre jugement sur la mesure qui nous est proposée. Nous sommes bien en présence de ce que l'économiste Gabriel Zucman qualifie de « bombe à retardement » pour les finances publiques et que, pour ma part, je nommerai sans hésitation une forme d'« évasion fiscale légale ». L'étude de l'OFCE, publiée au mois de juin dernier et affinée depuis, apporte les précisions suivantes, une fois appliqué au dispositif le modèle macroéconomique de l'Observatoire en matière de fiscalité et de distribution des revenus : « Selon nos Selon nos simulations, réalisées à l'aide du modèle de microsimulation Ines, développé par la DREES et l'INSEE, le " PFU à 30 % ", avec la liberté laissée aux contribuables de choisir le mode d'imposition le moins élevé, devrait impacter positivement environ 12,8 millions de ménages pour un coût budgétaire de l'ordre de 4 milliards d'euros, soit un gain moyen de l'ordre de 315 euros par ménage bénéficiaire. Si seuls 16 % des ménages du premier décile de niveau de vie voyaient, à la suite de la réforme, leur imposition sur les revenus mobiliers décroître,

d'abord sur les flux, ensuite sur le stock. La fiscalité du capital n'est pas assez aux services de la croissance : elle n'incite pas les entreprises à investir et pénalise notre pays par rapport à ses voisins.

Évidemment- nous aurons l'occasion d'en reparler -, notre système fiscal est biaisé en faveur de l'immobilier. Je sais que cela suscite des débats, mais, dans ce cas-là, il faut prévenir toutes les personnes qui investissent dans l'immobilier et qui sont si attachées à la pierre. D'ailleurs, de ce point

Ce n'est pas le seul problème soulevé par cette mesure. Elle est en effet particulièrement inégalitaire. Avec le PFU, qu'il faut replacer dans la logique de la suppression de l'ISF, les cent premiers contribuables à l'ISF gagneront chacun, en moyenne, environ 1,5 million d'euros par an. De plus, le bénéfice lié à la mise en place du PFU est extrêmement concentré : 44 % du gain total est capté par le 1 % des ménages les plus aisés. Je ne reviendrai pas sur la démonstration de l'économiste

la mesure où il pourrait y avoir de l'optimisation fiscale, cette mesure pourrait faire perdre à l'État plus de 10 milliards d'euros par an. En effet, la permettra à certains de se payer sous forme de dividendes, sans acquitter les prélèvements sociaux, ce qui entraînera un fort manque à gagner pour le budget de la sécurité sociale et le budget Des dispositions fiscales similaires appliquées par d'autres pays, comme la Finlande ou les États-Unis, ont ainsi montré que ces mesures favorisaient l'optimisation fiscale. Par ailleurs, tout comme l'article 12 qui remplace l'ISF par l'IFI, l'article 11 offre un avantage fiscal substantiel aux contribuables les plus riches, alors que, dans le même temps, les plans d'épargne logement,

je souhaite, au début de notre débat sur un point majeur du projet de loi de finances pour 2018, expliquer le sens du choix politique fait par le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du Gouvernement. Instaurer un prélèvement forfaitaire unique sur les intérêts du capital, c'est un gage de simplicité dans un dispositif fiscal aujourd'hui mité par les exceptions et règles particulières, qui empêchent de donner de la lisibilité à l'épargne. C'est également un gage d'efficacité, parce que notre économie a besoin d'être mieux financée. Face à des révolutions technologiques qui sont de plus en plus rapides, le besoin en capital va être de plus en plus important. L'alternative est très simple : soit nous continuons à taxer le capital au niveau où il est aujourd'hui et nos entreprises ne pourront pas financer les investissements nécessaires et leur modernisation, soit nous

va vers des placements sûrs plutôt que vers l'économie et les entreprises. Nous proposons de rompre avec ce système-là pour aller vers un système fiscal plus favorable au financement de notre économie.

l'analyse faite par M. Zucman, qui est sans doute très fondée pour l'économie américaine, mais l'est beaucoup moins pour l'économie française et les entreprises françaises. Quant à l'analyse de l'OFCE, elle a été réalisée avant que le dispositif PFU soit précisé. ne tient notamment pas compte du fait que nous avons choisi de soumettre au prélèvement forfaitaire unique l'ensemble des contrats d'assurance vie dont l'encours est supérieur à 150 000 euros.

I-221. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, 749 163 : c'est le nombre de ceux qui ont quelque intérêt à voir s'appliquer l'article 11 que le Gouvernement entend soumettre à la décision du Parlement.

Par rapport à la réforme de la taxe d'habitation, les choses sont plus simples. L'État est censé perdre environ 1,3 milliard d'euros en 2018 et aux alentours de 1,9 milliard d'euros les années suivantes. se pose -sera payée par les autres contribuables, qui perdront en réduction de la dépense publique ce que d'autres pourront garder par-devers eux, avant de se mettre à l'affût d'un nouveau juteux placement de leurs petites économies. Pour reprendre un exemple que nous avons évoqué lors du débat sur la taxe d'habitation, l'article 11 intéresse par exemple environ 8 000 familles de Neuilly-sur-Seine qui disposent de plus de 2,4 milliards d'euros de revenus et paient 615 millions d'euros d'impôt sur le revenu. À Loos, dans ma région, dans la banlieue lilloise, 57 contribuables ont déclaré plus de 100 000 euros, pour un montant global de 9,4 millions d'euros et un peu moins de 2 millions d'euros d'impôt à payer. Ces données simples montrent les enjeux et illustrent clairement l'objectif du dispositif. Pourquoi faire référence à ce seuil de 100 000 euros ? Tout simplement parce que, selon les éléments fournis par les sites du ministère, ce n'est qu'à partir de ce seuil d'imposition que le taux apparent d'imposition excède les 12,8 % forfaitaires. Eh oui, les seuls contribuables ayant un quelconque intérêt à voir s'appliquer l'article 11 ne peuvent être, par principe, que ceux dont le revenu global est soumis à un prélèvement supérieur à 12,8 Les retraités, prévenants pour leurs petits-enfants, qui mettent quelques sous de côté au guichet de leur banque de dépôt n'ont strictement aucun intérêt à passer par le régime de l'article 11. Pour ne rien arranger et, probablement pour pousser à l'achat des stocks de logements invendus de quelques dispositifs d'investissement immobilier incitatifs,

d'une importance vitale pour la France. Vous auriez trouvé là une enveloppe qui aurait directement financé l'entreprise française sans passer par les actionnaires. Enfin, cette

extrêmement complexe, avec des taux différents- on en a détecté plus de quinze sur les gains de cession en capital -, ce qui rend le système illisible. L'une des convictions de la commission, c'est que l'acceptation de l'impôt passe sa lisibilité, par des bases fiscales larges et des taux les plus faibles possible.

le risque d'érosion de la base ou de transfert d'une partie des revenus, notamment de dirigeants qui sortiraient du barème et préféreraient aller vers le prélèvement forfaitaire unique, privilégiant le paiement en dividendes plutôt qu'en salaires.

dans un second temps, c'est-à-dire l'année prochaine, de réfléchir à des dispositifs permettant de mieux associer les salariés aux résultats de l'entreprise. Le Président de la République l'a dit- tous les gaullistes qui sont présents dans cette enceinte, et ils sont très nombreux, y sont attachés autant que moi -, l'objectif est que, à terme, 100 % des salariés aient accès à un dispositif d'intéressement ou de participation,

il n'y ait pas que les actionnaires qui en profitent, mais que les salariés, qui sont la première richesse des entreprises, en bénéficient aussi. Ne limitons pas le raisonnement du Gouvernement à la seule amélioration des marges et des profits des entreprises. Nous le faisons avec, en perspective,

Tout cela n'est pas suffisant et n'a pas encore un impact suffisamment fort sur le chômage. J'ai fixé à deux ans le moment où nous pourrons juger des effets de cette politique sur le redressement de l'emploi dans notre pays : le redressement sur le fond prendra plus de temps et ne se fera pas du jour au lendemain. C'est justement parce que cela va mieux et que les perspectives de croissance en France, en Europe et dans le monde sont positives que c'est le bon moment pour mettre en place ce prélèvement forfaitaire unique.

Cet amendement vise à maintenir l'imposition au taux de 30 % des gains réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, les BSPCE, lorsque le contribuable exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution de ces bons depuis moins de trois ans. Il s'agit de revenir au régime antérieur, le régime fixé aujourd'hui étant défavorable.

les socialistes ont toujours combattu cette idée, ils lui trouvent soudainement beaucoup de qualités lorsqu'il s'agit de contester une mesure gouvernementale qui, par ailleurs, peut effectivement être critiquée ou amendée.

indépendants, le bénéfice du prélèvement forfaitaire unique serait plafonné à la part du revenu n'excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d'associé. Là encore, une telle mesure trouve son inspiration

les sociétés au profit des travailleurs indépendants sont soumises aux cotisations du régime social des indépendants pour la part dépassant 10 % du capital social et du compte courant d'associé.

matin. Ce prélèvement à la source s'accompagnera d'un effacement de l'impôt sur les traitements et salaires perçus en 2018, alors que les dividendes, eux, seront soumis au prélèvement forfaitaire unique.

positive, nous restons tout à fait défavorables au principe même du prélèvement forfaitaire unique, ainsi que l'a fort justement souhaitez accroître la profitabilité des entreprises, c'est votre credo, mais vous le faites au prix de la détérioration de nombreux services publics. Ainsi, vous améliorez le capital de ceux qui en ont

Nous sommes aussi attachés que vous aux services publics, nous sommes aussi attachés que vous à la redistribution, nous sommes aussi attachés que vous à la bonne rémunération des salariés, ... Et des fonctionnaires entre vous et nous, c'est que vous pensez qu'on peut redistribuer des richesses avant de les avoir créées. Voilà ! Nous, nous estimons qu'il faut d'abord créer des richesses avant de les redistribuer. C'est le b.a.-ba ! Je suis désolé de le souligner, mais si la France s'est appauvrie depuis des années et des années, c'est parce qu'elle n'a cessé de redistribuer des richesses qu'elle n'avait pas créées. Nous avons voulu financer des services publics alors que nous n'avions pas l'argent pour cela. Bien sûr ! Nous avons voulu aider ceux qui en avaient le plus besoin sans en avoir les moyens.

que si nous ne taxons pas demain les données, qui sont les principales créatrices de valeur, nous n'aurons pas de quoi financer nos services publics, nos crèches nous hôpitaux, nos écoles. préoccupations : bien financer nos services publics, aider les plus fragiles, mais il y a une différence absolument majeure entre vous et nous, je le répète, c'est que vous pensez qu'on peut le faire sans créer de richesses, quand nous pensons qu'on ne pourra le faire, et continuer à le faire, qu'en créant plus de richesses.

prévoyez que l'abattement proportionnel maintenu pour les cessions de titres acquis ou souscrits avant le 1 janvier 2018 puisse auparavant se cumuler avec l'ancien abattement fixe de 500 000 euros. Vous rétablissez la possibilité d'un cumul, plus le PFU, ce qui constituerait un double avantage. Pour cette raison, le

avec cet article 11, nous allons procéder à la réduction de la fiscalité pesant sur les revenus du capital, puisque la plupart des produits financiers existants échapperont à l'application du barème progressif. Un dividende de 100 000 euros nets de CSG taxé à 12,8 %, c'est tout de même nettement mieux qu'à 45 %, puisque cela fait 32 200 euros de plus pour le détenteur sans doute bien plus que ce que représente la prime accordée aux détenteurs de comptes ou de plans d'épargne logement, qui vont devoir s'acquitter demain du prélèvement forfaitaire unique,

Le fait est que l'article 11 élargit l'assiette du PFU à quelque chose comme 262 milliards d'euros, à fin mars 2017. On se demande bien pourquoi cette somme n'est pas mobilisée pour financer plus directement l'économie. Comme si les établissements qui collectent cette épargne grassement rémunérée à 0,50 % n'en faisaient rien

Entre la rémunération de l'épargne logement, qui sert tout de même d'apport personnel pour nombre de familles accédant à la propriété d'une maison ou d'un appartement, et les taux offerts sur le marché, il y a encore de la marge. À partir du 1 janvier, cette épargne va donc être taxée, ou plus précisément les intérêts qu'elle dégage, ce qui fera, pour l'an prochain, si rien ne change, environ 1,3 milliard d'euros d'intérêts taxables, soit 390 millions d'euros

il n'est pas rare que, dans cet hémicycle, de droite à gauche en passant par le centre, on trouve des points de convergence. Il est vrai que c'est un peu dans la nature du Sénat. En ce qui concerne les plans d'épargne logement, vous l'avez compris, monsieur le ministre, demandons le respect d'une forme de logique, notamment pour éviter la brutalité d'une mise en oeuvre de la nouvelle mesure à partir du 1 janvier et puis pour fiscaliser les intérêts. Tel est

j'attire en même temps l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre en compte, dans le parcours résidentiel

moins favorables, à la fois en taux et en durée, pour les ménages qui veulent acquérir une propriété. Il faut absolument retravailler pour proposer de nouveaux dispositifs

pour les ménages, quel que soit leur niveau de ressources. Hier, nous avons eu l'occasion d'évoquer notamment toute la problématique du logement locatif. On voit que, dans la panoplie, entre le locatif et l'accession à la propriété,

présenter l'amendement n° I-129 rectifié. Le présent amendement vise à rapprocher en 2022 le taux du PFU, prélèvements sociaux inclus, de celui en vigueur chez nos principaux voisins européens, notamment en Italie et en Allemagne, où il est de 26 %, en réduisant le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu de 12,8 % à 8,8 %.

Comme vous le savez, les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés vont être soumises à un prélèvement forfaitaire au même taux que les revenus du capital tels que les dividendes ou les intérêts, sans prise en compte de la durée de détention. Une telle absence soumet donc au même régime les plus-values spéculatives de court terme et celles résultant d'une accumulation de valeurs sur plusieurs années, comme c'est le cas notamment de celles qui sont réalisées par les actionnaires des entreprises familiales. Pour prendre en compte ces situations et favoriser l'investissement de long terme, le présent amendement vise à réduire le taux de prélèvement forfaitaire à 5,8 % lorsque les actions ont été détenues pendant au moins cinq

qui nous divisent Je comprends le souci du président de la commission des finances, mais je voudrais attirer son attention sur le fait que le Gouvernement

Si nous commençons dès maintenant à figer dans le marbre les critères d'évaluation de la politique fiscale, alors même que nous allons confier à des parlementaires, à des fonctionnaires à des responsables d'organismes indépendants le soin d'évaluer cette politique fiscale, j'ai peur que nous ne limitions l'efficacité du dispositif. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Ainsi, bien que je partage totalement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

prévoit, très concrètement, de ramener le taux d'imposition de ces plus-values à hauteur de 12,8 % au lieu de 16 %, sans doute en vue de « neutraliser » les effets de la hausse de la CSG. Une CSG portée à 17,2 % enfoncerait en effet un coin de 33,2 % de prélèvements sociaux et fiscaux dans le total de la plus-value encaissée Une situation à vous décourager de vendre un immeuble ou de céder quelques actions détenues de long terme et peut-être de famille. On nous dit qu'il s'agit en fait de rétablir l'équité entre les détenteurs de capitaux. Ainsi, en plus d'être une bombe à retardement, le prélèvement forfaitaire unique est aussi une sorte de bombe à fragmentation, si je puis me permettre l'expression. Nous rappellerons juste à nos gouvernants que le code général des impôts traite, au travers de plusieurs articles, de la question des plus-values. L'article 151 fixe, entre autres choses, un plafond d'exonération, qui atteint tout de même la somme de 250 000 euros de recettes constatées pour une activité de vente de marchandises en magasin. De son côté, l'article 39 permet d'imputer les plus-values sur les déficits constatés. Autant dire que nos collègues députés ont voté une mesure qui ne trouvera pas tant que cela à s'appliquer et dont l'impact sera fortement limité. Accessoirement, la valeur d'une entreprise n'est pas toujours liée au seul talent de son responsable, aussi grand soit-il. N'oublions pas les salariés, qui sont eux aussi

général, de porter l'abattement prévu en cas de donation à des petits-enfants de 31 865 euros à 70 000 euros. L'idée de pouvoir transmettre plus facilement, en franchise d'impôt, me paraît une idée louable, que je peux parfaitement comprendre. Pour autant, je rappelle que le montant d'abattement que nous avons prévu est déjà

si l'on cumule l'ensemble des abattements applicables. Je rappelle enfin que l'ensemble du coût de cette mesure d'abattement est déjà de 180 millions d'euros pour le

! Le Gouvernement souhaite effectivement favoriser le financement en actions de notre économie, mais je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'ouvrir l'accès au PEA dès l'âge de 16 ans. Nous préférons maintenir l'âge

que nous demanderons soit aux banques soit aux assureurs de mettre en place pour que le capital libéré aille effectivement vers le financement de l'économie réelle, notamment vers les PME. Pour autant, ces évolutions ne me semblent pas passer par un PEA ouvert dès l'âge de 16 ans.

un patrimoine que j'appellerai moins risqué que celui que l'on peut constituer avec des titres ou des parts de sociétés et que nous avons vu se développer, au fil du temps, notamment en raison de sa rentabilité. La loi de décembre 1948 avait donné un coup d'arrêt à certaines formes de spéculation immobilière, ... Et organisé la pénurie de la loi Méhaignerie de décembre 1986 a sensiblement relancée. Ont notamment été adoptées des mesures phares comme la libération des loyers du secteur privé- forte consommatrice d'aides au logement -et la mise en place du congé-vente, qui a engendré les copropriétés dégradées qui continuent de marquer le paysage de nos centres-villes anciens ou de certaines communes de banlieue. J'y ajoute l'amendement dit Marini sur le statut des foncières, qui a favorisé les ventes à la découpe et renforcé les antagonismes et la concurrence sur le marché immobilier entre les propriétaires bailleurs dits physiques et les investisseurs immobiliers institutionnels. Là est, à notre avis, le débat qui nous occupe en arrière-plan de cet article 12. La création de l'impôt sur la fortune immobilière,

Or les conventions fiscales avec le Qatar et un certain nombre d'autres pays du Golfe exonèrent les plus-values immobilières et les revenus immobiliers des résidents de ces pays.

de succès, puisque le nombre de contribuables qui ont sollicité son application est faible. Son coût s'élève pourtant à 190 millions d'euros pour les finances publiques. La même remarque vaut pour la disparition du régime ISF-PME, qui n'a plus de raison d'être. Cet article est une incitation marquée à l'instabilité actionnariale, aux placements de circonstance fondés sur l'espérance d'une plus-value rapide, c'est-à-dire exactement tout le contraire, me semble-t-il, de ce qu'il conviendrait de faire pour stabiliser le capital de nos PME. cela est coûteux pour les finances publiques, injuste du point de vue de l'égalité devant l'impôt- l'ISF est une bonne illustration de la capacité contributive des plus aisés -et, enfin, inefficace sur un plan économique, puisque cela va fragiliser les noyaux d'actionnaires de moult PME de notre pays. Cet article qui

c'était le terme employé en 1982. Aujourd'hui, c'est l'ISF, et il ne s'agit pas juste d'un changement sémantique. En effet, aujourd'hui, cet impôt, du fait des évolutions de patrimoine, est de moins en moins un impôt sur les grandes fortunes, et de plus en plus un impôt sur les petites fortunes. Tout à fait ! Les grandes fortunes,

qu'investir en bitcoins est plus bénéfique pour l'économie que d'investir en appartements ? Est-ce qu'investir

pour d'autres raisons, que j'ai exprimées à l'instant. En revanche, défendre l'IFI est vraiment la plus mauvaise solution. Vous auriez créé un impôt sur la fortune improductive, on aurait sans doute pu vous suivre. Si vous aviez réintégré les liquidités, tout ce qui est improductif,

je partage une partie de vos propos et, vous le savez, le Gouvernement également. En même temps, en ce qui me concerne, j'ai une règle assez simple : quand, comme ministre en charge des relations avec le Parlement, je dois accompagner la mise en oeuvre d'un engagement

l'ISF permet de régler les problèmes de pauvreté que nous connaissons en France. Si cela était vrai, peut-être ne serions-nous pas seulement l'un des trois pays européens à avoir ce type de fiscalité, qui a depuis longtemps montré son inefficacité, et qui a poussé de a poussé de nombreuses personnes à jouer soit de l'optimisation fiscale, soit de la fraude fiscale, soit, même, du déplacement physique pour quitter la France et échapper en totalité à la fiscalité et aux impôts sociaux. On sait donc l'inefficacité de ce dispositif. C'est simple, si cela marchait, cela se serait vu, et les recettes fiscales de notre pays se porteraient mieux. Surtout, d'autres pays européens auraient pu s'en inspirer, or je vous rappelle que seules l'Espagne et la Norvège ont aujourd'hui un dispositif qui se rapproche. Il y a la Suisse, mais mais je ne suis pas sûr que le modèle fiscal de la Suisse soit celui que nous souhaitions tous partager ici. Cela montre bien la limite de cet argument qui consiste à dire : ne changeons rien ! D'autre part, il y a une vision plus ambitieuse,

je dis toute l'économie, c'est aussi la détention d'une PME, y compris la possibilité de transmettre à son fils ou à sa fille, un jour, l'entreprise familiale. C'est un élément très important qui est traité par l'article que vous proposez de supprimer.

L'accumulation de détention de capital immobilier ne contribue pas à la richesse nationale. On peut imaginer aujourd'hui de garder le système tel qu'il est. Je vous rappelle que, sur l'immobilier, nous n'augmentons pas les taux et nous ne diminuons pas l'assiette. Pour nous, il est indispensable de considérer qu'un meilleur partage de

vous avez besoin d'investisseurs privés et publics, et vous mettez les bailleurs sociaux en difficulté. Effectivement. Vous rendez-vous compte de l'ensemble des signaux que vous envoyez ? Or nous vivons une crise du logement et nous avons besoin de construire. Quand le bâtiment va, tout va,

les sondages ne vous condamnent si vous aviez supprimé totalement l'ISF ? Eh oui ! Mais quel est le risque que vous prenez en maintenant cet impôt uniquement sur l'immobilier, plus tout le reste, dont nous parlerons au moment de l'examen de l'article 52 ? Si, effectivement, c'est pour replanter le marché de l'immobilier, alors qu'il est reparti très fort à la hausse après le creux des années post-Duflot,

Je reconnais bien que nous n'avons pas eu le courage, sous les gouvernements de droite, du temps de Sarkozy, par exemple, de supprimer l'ISF, alors qu'une grande partie de nos troupes condamnait cet impôt. Nous n'avons pas eu ce courage, et je reconnais bien volontiers que le Gouvernement a le courage, lui, de prendre une décision que nous n'avons pas prise. Seulement, on a le sentiment que vous ne voulez pas aller au bout.

veulent acquérir leur logement pour leur retraite ; c'est un acte de confiance, c'est quelque chose qui les rassure. Il ne s'agit pas de capital dormant : c'est tout simplement de la prévision. Autrefois, on recommandait d'économiser pendant

Trouvons des solutions plus équilibrées, qui jouent à la fois sur la réduction des dépenses de l'État et la fiscalité sur l'activité, mais, par pitié, n'assommez pas l'immobilier.

collègues, tout a été dit par notre groupe : nous considérons que l'ISF est un impôt qui ne paralyse pas l'économie nationale et qui contribue à une certaine justice sociale. Non, il ne paralyse pas l'économie nationale

avez une vision dogmatique, selon laquelle plus on allégera les riches, quelles que soient les formes de leur richesse, plus l'économie se portera bien. Cela n'a jamais été prouvé

Entre la rente foncière et la pseudo-rente immobilière de tous les secteurs de l'immobilier, on ne peut pas faire un tout homogène. Nous n'avons pas

on demande des efforts sur le travail, sur les emplois aidés, sur les contrats aidés ; on demande des efforts sur le logement et on sait l'impact que cela aura ; on demande des efforts aux collectivités. En même temps, on enlève ces 5 milliards d'euros des recettes de l'État : c'est ça qui ne va pas.

qui est un impôt confiscatoire, totalement inutile, stupide, qui frappe particulièrement les millionnaires, qui a fait fuir les milliardaires.

En revanche, je ne suis pas l'analyse de mes collègues de droite, et je voudrais saluer le courage de ce gouvernement. Il faut être cohérent et constant dans nos opinions. Un septennat et un quinquennat de Jacques Chirac n'ont pas permis de supprimer l'ISF ; un quinquennat de Nicolas Sarkozy n'a pas permis de supprimer l'ISF pour la première fois, un gouvernement se penche sur la question et propose de supprimer les trois quarts de l'ISF. Nous ne pouvons pas ne pas saluer cette initiative. J'entends dire

C'est la raison pour laquelle, face à une difficulté de choix, et voulant saluer la démarche du Gouvernement, les Indépendants, même s'ils sont hostiles à l'ISF,

de cette polarisation de la fiscalité sur ce secteur économique, en ayant bien en tête que Bercy -il faut toujours dire que cela vient de Bercy ; Bercy a bon dos -considère que, l'activité économique étant suffisamment bonne aujourd'hui,

finirez par noyer la cause que vous prétendez défendre. Je crois donc qu'il y a un sujet, et le Sénat est là pour attirer l'attention sur le besoin de corriger le système nouveau que vous entendez mettre en place, même s'il faut vous donner acte du courage de supprimer l'ISF.

je préfère être rapide. Monsieur le ministre, nous comprenons très bien votre volonté d'avancer sur le sujet. Nous la saluons, bien sûr, elle a d'ailleurs été saluée par mon groupe.

Et il me semble que l'un des maux dont souffre aujourd'hui l'agriculture, c'est l'absence d'investisseurs. Expliquez-moi pourquoi le fait d'investir dans du foncier agricole, ce serait investir dans de l'économie irréelle ou dans de l'économie qui n'existerait pas.

Ce que je constate, c'est que l'immobilier, par définition, ne se délocalise pas. Voilà ! Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez jeter l'anathème sur l'immobilier ! La deuxième réflexion que je voudrais faire est d'ordre purement sémantique.

soutenu. Reprenant les propos de notre collègue Philippe Dallier, je voudrais rebondir sur l'image que ce gouvernement donne de l'immobilier. On a parlé bien évidemment du logement.

effet, nous vivons un choc économique, avec la répartition mondiale des activités et la nouvelle organisation des entreprises. Nous vivons un choc technologique, avec la numérisation.

l'économie, c'est aussi une affaire de signal, notamment pour renforcer l'attractivité. C'est une affaire de dynamique. Et cette réforme engage une dynamique. Sur l'immobilier,

Au contraire, le goût pour la pierre, la volonté d'investir dans l'immobilier, que ce soit en France ou à l'étranger, sont encore très puissants dans notre pays. Il faut donc aussi

d'abord, que je trouve le Gouvernement courageux de supprimer la partie mobilière de l'ISF. Je voudrais simplement rappeler à nos collègues de droite que nous avons appartenu, les uns et les autres, à une majorité qui l'avait tout autant supprimée.

lutter contre de vraies rentes immobilières, celles qu'autorise la puissance publique lorsqu'elle donne à des propriétaires fonciers des avantages tels qu'ils

battons-nous sur les normes, battons-nous sur la constructibilité et bien évidemment sur l'apport de capitaux pour construire ces logements dont nous avons besoin ! Vous ne tiendrez pas deux ans avec votre impôt sur la fortune immobilière, parce qu'on a besoin d'argent dans l'immobilier pour répondre aux besoins de nos compatriotes

secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne répondrai pas à toutes les questions, mais je voudrais vous rassurer. D'abord, il n'y a aucune raison de laisser penser à celles et ceux qui veulent investir dans l'immobilier qu'une fiscalité nouvelle, punitive, changerait la donne. Nous ne changeons rien

le propriétaire n'est pas l'exploitant, il bénéficie d'une détaxe particulière à 75 %, et donc, là encore, il n'est pas impacté par l'ISF. Je crois donc que l'agriculture n'est pas forcément le meilleur exemple. En effet, dans 98 % des cas, le producteur d'économie réelle, l'agriculteur- et je suis d'accord avec vous, il produit, il est dans l'économie réelle, une salade est une forme d'économie réelle -est exonéré en exonéré en totalité du fait de la détention de son patrimoine immobilier. Je pense que c'est important. Monsieur le rapporteur général, vous avez relevé quelques anomalies

deux éléments au débat en cours. On entend parler d'exode. L'ISF ferait fuir les fortunes ... Je n'ai pas les chiffres les plus récents, j'ai les chiffres de 2014. 784 foyers concernés par l'ISF qui auraient quitté le territoire quand 300 rentraient sur le territoire. Cela fait donc un solde négatif de 484 sur 330 000 foyers

là, l'ISF est un impôt stupide, idiot ... ! On peut toujours justifier la suppression d'impôts qui dérangent quelque part. L'impôt intelligent, à mon avis, c'est un impôt juste, progressif et auquel personne n'échappe. Second élément que je livre à la réflexion de chacun je vous renvoie au discours de Mme Christine Lagarde, qui n'a pas pris sa carte au parti communiste, ... Pas encore ! ... je vous rassure, en tout cas, je n'en suis pas informé. C'était à Harvard, le 4 octobre 2017, Mme Lagarde faisait la promotion d'une hausse des impôts pour les plus riches ... Elle s'en partant du constat objectif que les inégalités excessives pénalisent la croissance. Quelle belle idée ! On devrait y réfléchir

placé en bons du Trésor américain, c'est productif pour l'économie réelle », peut-être, moi, j'ai quelques doutes. En revanche, je suis certain qu'avoir des terres agricoles avec des agriculteurs pour les exploiter, cela contribue à l'économie réelle. le fait de posséder des appartements, des biens immobiliers qui sont loués et qui servent à loger des personnes- je vous rappelle qu'un quart des foyers français sont logés dans le secteur locatif privé, à 98 % détenu par des personnes physiques cela contribue à l'économie réelle. Posséder une usine, un entrepôt, cela contribue à l'économie réelle. Donc, je ne comprends pas la logique qui consiste à centrer cet impôt exclusivement sur l'immobilier et à laisser de côté tout ce qui est totalement improductif, y compris les pires horreurs ! Je parlais des bitcoins, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Si vous aviez créé un impôt incluant dans son assiette les liquidités, les placements de pur plaisir, les résidences secondaires, sur lesquels il n'y a pas de justification particulière à la contribution à l'économie réelle, on aurait pu avoir une assiette, puisque vous avez besoin d'un rendement, à peu près 850 millions d'euros. Vous avez fait le choix de vous concentrer exclusivement sur l'immobilier, peut-être

est exclu du PFU, il reste soumis au barème de l'IFI, les mesures de l'article 52, la concentration sur la taxe foncière, le prélèvement à la source, qui l'année prochaine, s'il était mis en oeuvre, diminuerait la possibilité de déduction des travaux, etc. Il y a malheureusement une convergence de toutes les mesures fiscales qui vont à l'encontre de l'immobilier à un moment où les Français ont besoin de se loger. Pour éviter à la présidente de me couper la parole, de me rasseoir et de redemander la parole, je finis mon propos. Je dis simplement que l'impôt tel qu'il est conçu est une très mauvaise idée. Il aurait mieux valu, à la rigueur, créer un impôt sur la fortune immobilière, on aurait pu vous suivre, on aurait pu éventuellement en discuter, mais vous avez fait le choix de l'immobilier. Il risque d'avoir des effets pervers. En plus, vous avez fait le choix de la complexité parce que vous êtes allé chercher les actifs, et ce sera très compliqué. Je le dis solennellement à tous les collègues qui n'ont pas eu le temps d'étudier le dossier, l'IFI est beaucoup plus compliqué que l'ISF parce qu'il faudra regarder dans chaque placement,

Or dans les faits, l'ISF est aujourd'hui insuffisant- je n'ai pas dit inutile -pour répondre à ces deux exigences. L'assiette de cet impôt est largement tronquée puisque nombre de biens parfaitement représentatifs de la réalité des patrimoines les plus importants sont exonérés ou pris en compte très en deçà de leur valeur. Quant à son taux, il n'a jamais été une source de difficulté majeure pour les contribuables assujettis. Cet amendement a donc pour objet de revenir au principe de réalité en faisant en sorte que la justice la plus élémentaire s'applique entre les contribuables. Nous n'avons jamais jugé normal- et j'insiste sur ce point -que les biens professionnels se trouvent exclus de l'assiette de l'ISF, d'autant qu'il ne s'agit bien souvent que de titres et de parts de sociétés, un patrimoine dont la matérialité se résume à celle de morceaux de papier imprimés. Ainsi, persiste dans notre fiscalité un traitement différencié des titres, à nos yeux injustifié : exonération de droits pour les biens professionnels, exonération possible en cas de participation à un pacte d'actionnaires qui, en règle générale, n'entraîne d'ailleurs aucune conséquence en termes d'implication desdits actionnaires dans la vie quotidienne de l'entreprise concernée, exonération impossible pour les titres détenus par des actionnaires minoritaires n'étant pas liés par un tel pacte. Notre démarche est simple : rendons imposables les biens professionnels au-delà du seuil de 2 millions d'euros afin de rétablir l'égalité de traitement entre les actionnaires

que vous n'avez pas tenu compte du fait que l'année prochaine on pourra imputer l'ISF-PME qui continuera. Monsieur le secrétaire d'État, je vous pose une question précise : les 850 millions d'euros de rendement attendus et annoncés tiennent-ils compte du fait que, l'année prochaine, on pourra encore bénéficier de la réduction ISF-PME ?

comptable des engagements présidentiels. Car ce dont nous parlons était effectivement au coeur de l'engagement présidentiel. Il ne s'agit pas de baisser l'impôt pour baisser l'impôt. Il ne s'agit pas de dire qu'on veut moins de recettes fiscales. Il s'agit d'encourager l'investissement

le rappelle, à partir d'un certain niveau, 1,3 million d'euros de détention de patrimoine qui engendre le premier niveau de taxation sur l'ISF et seulement à cette échelle et à ce niveau. Cela signifie qu'au fond nous encourageons les détenteurs de patrimoine à prendre un risque.

celui de tout perdre, ce qui n'est pas le cas en matière immobilière et c'est là le pari ! Au fond, il n'y a pas de désaccord sur ce sujet entre nous. Vous avez une ambition fiscale. Nous avons une ambition d'orientation d'investissements vers l'économie, vers l'économie productive et, donc, vers l'emploi. C'est là que se situe la différence. Oui, on pourrait imaginer- et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous -de flécher un certain nombre d'investissements qui ne seraient pas assez productifs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, par exemple, sur les liquidités qu'on laisse dans un compte en banque. En effet, l'économie bancaire contribue à financer l'économie réelle ... Comme

Nous n'avions pas voulu l'inscrire parce que nous voulions la simplicité entre deux blocs, le bloc d'investissement et le bloc de détention de patrimoine. Les parlementaires, les députés- encore eux

l'objectif, c'est quelque chose de simple. Et le dispositif qui vous est proposé est relativement simple. N'oublions pas de quoi on parle ! Je voudrais rebondir sur l'ISF belge. Oui, la Belgique fait le choix d'instituer un taux d'ISF qui, pour 500 000 euros de détention, va engendrer 750 euros de recettes.

l'impact sur le rendement de l'IFI de l'imputation de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés avant le 31 décembre 2017 n'a pu être estimé ». L'année dernière, la réduction ISF-PME représentait 660 millions d'euros.

d'un certain nombre d'exonérations particulières en ce qui concerne, en particulier, l'immobilier. J'aimerais avoir une réponse sur ce point : considérez-vous que les conventions fiscales actuelles continueront à s'appliquer,

deuxième remarque sur la rente immobilière : il faut comparer l'évolution des actifs. Or, à l'exception de rentes de situation auxquelles le pouvoir politique contribue parfois par des mesures de restriction,

ni demain dimanche, et nous pourrions reprendre l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances lundi matin, à dix heures.

-, ni de celui de la performance environnementale- impact environnemental des déplacements et des transports d'engins, consommation de carburant, gestion moins économe des traitements phytosanitaires

les incidences fiscales des échanges d'immeubles ruraux ne sont applicables qu'à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes. Cette limitation géographique est aujourd'hui difficilement justifiable et même paradoxale, dans la mesure où l'échange est particulièrement bénéfique s'il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d'une parcelle plus proche de son exploitation. C'est pourquoi nous vous proposons de supprimer la condition de proximité géographique pour l'application des dispositifs de faveur aux opérations d'échanges d'immeubles ruraux. En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. En effet,

proposons d'accorder une réduction d'impôt supérieure aux souscripteurs au capital des entreprises solidaires qui conservent leurs titres au moins sept ans. En effet, la suppression de la réduction ISF-PME, déjà évoquée, aura pour conséquence un recul important des investissements directs dans les entreprises solidaires. Rappelons que ces entreprises n'ont pas pour vocation de faire du profit. Elles offrent un faible rendement aux souscripteurs, ce qui ne permet pas d'attirer l'épargne privée. La réduction d'impôt est donc indispensable pour attirer des investisseurs au capital de ces entreprises et pour mobiliser des fonds propres

Notre amendement va dans ce sens, en prévoyant de maintenir un flux d'investissement direct dans les entreprises solidaires et en soutenant l'actionnariat solidaire, qui est un investissement citoyen, pérenne et efficace au service de la lutte contre l'exclusion sociale.

aurait une conséquence relativement grave : elle empêcherait le choc d'offre que nous voulons construire tous ensemble sur notre territoire et en particulier dans les zones tendues. Or c'est en Île-de-France, première des zones tendues, qu'aujourd'hui le foncier disponible et mis sur le marché ne permet pas d'atteindre des objectifs de construction de logements, qu'il s'agisse de logements sociaux, de programmes privés ou de toute autre forme juridique. Cette taxe aurait pour effet de renchérir le coût de l'immobilier justement dans les zones tendues, ce qui serait très négatif pour nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Le marché immobilier sur le territoire de l'Île-de-France est suffisamment difficile pour que nous évitions de rajouter un système de taxation qui pourrait pénaliser

à M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à exonérer complètement de la valeur des droits des biens retenus les transmissions familiales des exploitations agricoles.

aux contrats dits « article 83 » ou « loi Madelin », de prévoir le rachat, à partir de la cessation de l'activité professionnelle, de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats. Ces dispositions garantissent aux bénéficiaires qui partent à la retraite une hausse de pouvoir d'achat, tout en leur assurant des revenus réguliers viagers. elles ne prennent pas en compte la situation des affiliés des contrats retraite « article 83 », dont l'entreprise souscriptrice aurait disparu ou dont le contrat aurait été résilié. Dans ces cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne peut être proposé par l'assureur au souscripteur, puisqu'il n'y a plus d'entreprise. Il s'agit de mettre en situation d'égalité certains

le sénateur : le Gouvernement est défavorable à l'amendement, et il est prêt à être battu.

est à Mme Jacky Deromedi. Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l'étranger, de nombreux Français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leur pays d'accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.

de salaires avant impôt et que les fonds de croissance sont en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait. L'objet du présent amendement est d'inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l'impatriation fixé par l'article 115 B du code général des impôts.

sur les navires de plaisance, signe extérieur de richesse. Or c'est purement symbolique. D'après la Direction de la législation fiscale, cela ne devrait concerner que quelques unités ou quelques dizaines d'unités, pour une recette de moins de 10 millions d'euros. Il n'y a déjà pas beaucoup de grands

? Je ne connais pas de voitures françaises, achetées par des Français, de ce niveau-là de puissance, supérieur à 36 chevaux.

contribuer symboliquement et financièrement au redressement de nos comptes publics.

de taxer plus un certain nombre de véhicules, notamment les véhicules de plus de 15 chevaux fiscaux d'occasion. Il nous semble que

est à M. Éric Bocquet. L'impôt sur les sociétés est un impôt très largement corrigé par de multiples dispositifs tous plus coûteux les uns que les autres et grâce auxquels certaines entreprises paient un montant particulièrement faible d'impôt au regard de leur chiffre d'affaires réel et de leur résultat brut d'exploitation. En 2018, l'impôt sur les sociétés devrait dégager une recette nette de 28,4 milliards d'euros, largement entamée par le CICE notamment. Celui-ci va dépasser les 21 milliards d'euros et le crédit d'impôt recherche va ajouter 6 milliards d'euros à la facture des pertes de recettes. Le fascicule bleu « Évaluation des voies et moyens » nous indique que le régime d'intégration des groupes et le régime des sociétés mère-fille constituent des modalités particulières de calcul de l'impôt qui ont coûté 43,8 milliards d'euros de recettes fiscales en 2016. C'est cette situation problématique qui nous a amenés à déposer le présent amendement.

que les charges financières soient déductibles. Certes, depuis 2013, la déductibilité de ces charges a été très limitée, mais si l'on restreint encore cette possibilité, cela va être pénalisant pour les entreprises, particulièrement pour celles pour lesquelles vous supprimez les exceptions existantes. Je pense, par exemple, aux concessions de travaux publics. L'adoption de votre

tout en revenant sur la baisse uniforme du taux facial de l'impôt sur les sociétés jusqu'ici prévu. Rappelons à ce stade que nous avons, à l'article 2, proposé un barème de l'impôt sur le revenu qui avait la qualité essentielle de permettre aux travailleurs indépendants, eu égard à leurs revenus moyens, de disposer d'un allégement de leur fiscalité. nous nous occupons désormais de la question de nos PME, c'est-à-dire des entreprises dont le responsable principal est lui-même un salarié, en lieu et place d'un exploitant individuel. Comme chacun le sait, nous avons vu s'engager un processus de baisse du taux facial de l'impôt sur les sociétés qui pose d'incontestables questions. En effet, il y a belle lurette que la réalité de ce que perçoit l'État en bout de course n'a pas grand-chose à voir avec le taux affiché à l'origine. Quel est l'avis de la commission ? Quand nous

Cariou, avec un avis favorable du Gouvernement, et pour laquelle nous avons laissé passer ce qui pourrait paraître comme une coquille, mais qui, du fait de l'ajout d'une condition supplémentaire pour les sociétés établies dans l'Union européenne par rapport à celles qui le sont en France, pourrait formaliser une restriction de la liberté d'établissement, laquelle est garantie, je le rappelle, par le droit européen. Il s'agit de traiter de manière identique les situations, que la gestion de la participation soit exercée en France ou dans l'Union. Dans cet esprit, le présent amendement tend à supprimer l'exigence d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.